monsieur le président.

Nous votons toute une série de mesures liées à la crise du covid-19 qui prévoient des exonérations de cotisations sociales. La question du budget de la sécurité sociale va donc se poser avec acuité cet automne.

monsieur le ministre

le dispositif exceptionnel d'exonération de cotisations patronales, à l'aide au paiement des cotisations, aux remises de dettes et aux plans d'apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire du covid-19,

qui risque de le rendre peu incitatif dans un contexte où les contraintes spécifiques en outre-mer conduisent tous les observateurs à anticiper une haute saison touristique « morte Dans ce contexte, les entreprises n'auront pas d'autre choix que de recourir au chômage partiel et verront par ailleurs leurs charges fixes continuer à s'accroître.

En effet, nous estimons que le fait de prendre comme repère le revenu artistique de 2019 et imposer qu'il soit supérieur ou égal à 3 000 euros exclut un certain nombre de très jeunes artistes, notamment ceux qui ont débuté leur carrière

Toutefois, le plafonnement de cette dette sur une durée de trente-six mois apparaît comme insuffisant, notamment pour les entreprises en difficulté qui ont accumulé des dettes antérieures au 31 décembre 2019. Rappelez-vous les circonstances liées aux cyclones Irma et Maria.

de rehausser le plafond de l'étalement de la dette à soixante mois, à l'instar de ce qui avait été fait pour les plans Irma à Saint-Martin, sur appréciation de la CGSS locale. également de prévoir le premier paiement de l'échéancier au 31 janvier 2021. Enfin, nous proposons de prévoir une inscription au plan d'apurement de la dette par le cotisant et d'avancer la date de conclusion du plan d'apurement au 31 octobre 2020 au lieu du 31 décembre 2020, afin de permettre à certains cotisants de bénéficier de la dette sociale, ces derniers étant considérés, de fait, à jour de leurs cotisations.

se soucie des travailleurs indépendants affectés par la crise sanitaire et leur permet d'accéder à des dispositifs d'exonération de cotisations patronales, ainsi qu'à un plan d'apurement des dettes. Il faut se réjouir de ces mesures relativement novatrices. Toutefois, aucune mesure d'urgence n'est prévue par le Gouvernement pour les mandataires sociaux assimilés à des salariés du régime général de la sécurité sociale, qui sont dans une situation comparable aux travailleurs indépendants et dans une précarité tout aussi importante. Nous proposons d'étendre le bénéfice du dispositif prévu pour les travailleurs indépendants- exonération et plan d'apurement - aux mandataires sociaux assimilés aux salariés du régime général de la sécurité sociale listés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.

. La crise que nous traversons impacte gravement la santé économique des exploitations viticoles françaises. Le confinement et ses conséquences, mais aussi l'arrêt des exportations dû à la fermeture des frontières ont entraîné une sérieuse baisse des revenus de ces exploitations. Malheureusement, le calcul de leurs cotisations sociales est effectué sur la base des revenus passés, qu'il s'agisse de la moyenne des trois années précédentes ou de la seule année 2019. Ce calcul peut donc entraîner une importante distorsion entre le montant à régler et les recettes de l'année, impactées par la crise du covid-19. Pour éviter cette situation, nos collègues députés ont adopté un amendement visant à permettre aux exploitants ayant subi une perte de chiffre d'affaires de 50 au moins, entre le 15 mars et le 15 mai 2020, de calculer leurs cotisations sociales sur le résultat actuel, dit résultat de l'année N. C'est une avancée importante, mais elle laisse de nombreux agriculteurs de côté. C'est pour que cette possibilité soit élargie que nous proposons le présent amendement. L'amendement

L'impact négatif de la crise sur l'économie s'en trouvera aggravé, puisqu'il n'y aura pas d'activité compensatoire aux pertes enregistrées durant la période estivale à l'issue de celle-ci. Pour permettre aux entreprises de passer le cap difficile de l'exercice 2020, nous proposons une dérogation exceptionnelle-

Il s'agit du statut du personnel des GIP. Je me propose d'en rester là et de faire passer une note à M. le ministre, afin que celui-ci puisse apporter une réponse précise. Il faut néanmoins noter que certains de ces GIP, notamment des laboratoires, ont été fortement mobilisés pendant la période que nous venons de traverser.

à travers un dispositif d'exonération totale de charges patronales pour toute entreprise stratégique implantée à l'étranger qui déciderait de rapatrier sa production en créant des emplois en France. La liste des entreprises visées serait fixée par un décret en Conseil d'État.

de la transformation du CICE. Celle-ci concernait uniquement les cotisations d'assurance maladie pour les salaires inférieurs à 2,5 fois le SMIC. Quel est l'avis de

Il s'agit, non pas de reprendre le plafonnement existant dans les entreprises publiques- cela ne serait pas possible -, mais de fixer un écart type de 1 à 20

Cet amendement reprend la proposition de la Convention citoyenne pour le climat et vise à la rendre compatible avec la Constitution et le droit de l'Union européenne. Il s'agit d'augmenter la taxation des revenus distribués, c'est-à-dire les dividendes, les intérêts, les plus-values mobilières et les revenus d'assurance vie pour les primes, en la portant de 12,8 % à 16,8 %, lorsque le montant des dividendes perçus au cours d'une année dépasse un certain montant. Cette taxe frappe ainsi le récipiendaire du dividende, et non l'entreprise, mais l'esprit est le même que celui de la mesure portée par la Convention citoyenne. On le sait, cette proposition fait partie des jokers annoncés par le Président de la République, car elle est jugée décourageante pour les investisseurs.

Une telle taxation serait dans l'intérêt de tous. Un environnement sain, sans épisodes climatiques violents, une population en bonne santé, un climat social apaisé, cela nous semble être également dans l'intérêt des investisseurs. C'est en tout cas l'avis exprimé, en janvier 2020, par 121 millionnaires et milliardaires, qui appelaient leurs pairs à payer plus de taxes, estimant que les inégalités sont sources de violences sociales et que les impôts sont le seul moyen approprié pour assurer

contre 18 % pour un FIP finançant les entreprises continentales. L'économie insulaire, durement impactée par la crise, a besoin d'un apport d'investissements extérieurs pour soutenir l'activité. Porter à 50 % le taux actuel sur le seul exercice 2020 est de nature à favoriser l'investissement dans les entreprises insulaires, alors même qu'elles se trouvent particulièrement mises à mal, avec une structuration de l'économie reposant pour près d'un tiers sur le secteur touristique, qui subit de plein fouet les effets de la crise sanitaire, économique et sociale.

571 rectifié . Le déficit constaté au titre d'un exercice constitue une charge déductible du bénéfice réalisé au titre des exercices suivants. Toutefois, l'imputation du déficit sur l'exercice suivant est limitée à 1 million d'euros par an, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice supérieure à ce plafond. Cette règle de plafonnement du déficit reportable va conduire les entreprises à s'acquitter de l'impôt sur les sociétés dès qu'elles vont refaire des bénéfices, alors que leur situation sera encore très dégradée. collègues, de leur donner des marges de manoeuvre pour se relancer, en supprimant la limite d'imputation pour les déficits au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre, qui seront les plus impactés par la crise.

à Mme Jacky Deromedi. Le crédit d'impôt pour les investissements en Corse (CIIC) constitue depuis sa création un levier de développement des entreprises et de l'économie insulaire, trois fois prorogé par le législateur au gré des majorités parlementaires depuis 2002, tant son importance et son efficacité sont avérées. Arrivant à échéance au 31 décembre 2020, il est d'une impérieuse nécessité de le voir reconduit pour une période de cinq ans, et ce pour donner aux entreprises, dès à présent, de la visibilité sur un temps long afin qu'elles puissent envisager et réaliser sans attendre les investissements nécessaires à la relance ou à la poursuite de leur activité. La crise actuelle exige que l'on agisse au plus vite pour sécuriser le crédit d'impôt, alors même que l'économie corse se trouve fortement impactée et fragilisée.

il apparaît nécessaire de favoriser l'investissement dans les établissements de santé, par une politique fiscale incitative adaptée. L'article 244 E du code général des impôts, relatif au crédit d'impôt pour les investissements en Corse, concerne les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition et réalisant certains investissements productifs en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Néanmoins, les investissements éligibles sont limitativement énumérés, ce qui restreint considérablement la possibilité pour les établissements de santé d'en bénéficier. Le dispositif pourrait ainsi être élargi, afin de couvrir l'ensemble des investissements de ces établissements. Il est

considérant qu'ils ne peuvent y prétendre qu'au titre des « biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif » ou « des agencements et installations des locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle », contrairement aux hôtels, qui, eux, sont éligibles pour les travaux de construction et de rénovation. Alors que le secrétaire d'État de l'époque, Olivier Dussopt, avait considéré que l'amendement présenté dans le même sens lors du PLF pour 2019 n'avait pas lieu d'être, parce que satisfait par le droit en vigueur, l'administration fiscale infirme clairement cette position ... On va demander des noms ! ... et conclut de la façon suivante, dans un courrier du 15 mars 2019 :« Force est donc d'admettre que l'ensemble des investissements envisagés par les établissements de santé ne sont pas éligibles aux dispositions de faveur pour l'ensemble des investissements qu'ils entendent réaliser. Face à cette divergence de position persistante et au regard de l'intérêt de santé publique comme de l'urgence de la situation, la modification législative proposée par cet amendement est impérative pour permettre aux établissements de santé privés de bénéficier d'un levier indispensable pour répondre aux besoins de la population. Cet amendement, déposé à deux reprises l'an dernier, jugé à tort satisfait, est crucial afin de soutenir l'investissement dans les établissements de santé. La crise que nous traversons suffit à justifier le bien-fondé de cette précision légistique,

tout comme il convient d'encourager les entreprises à investir en 2021 pour garantir la relance de l'activité. C'est pourquoi le présent amendement vise à majorer de dix points le taux de crédit d'impôt, qui est de 20 % pour les PME et de 30 % pour les TPE. Quel est l'avis de

liées à l'implantation ou à la reprise d'activités en milieu rural, en ouvrant droit à des exonérations de fiscalité et à des allégements de cotisations patronales. Il s'agit donc d'un outil indispensable à la prise en compte des fragilités structurelles des territoires ruraux et au soutien direct à l'activité économique. Les mesures financières associées au classement en ZRR constituent en effet un soutien déterminant pour le développement des territoires. Cet outil, qui peut certainement être amélioré pour être rendu plus efficace, doit être pérennisé. Il joue un rôle essentiel pour aider les territoires à traverser la crise. Il est urgent de travailler dans de bonnes conditions à la révision du zonage annoncée par le Premier ministre lors de la présentation de l'agenda rural du Gouvernement. C'est un chantier important et complexe. La ministre de la cohésion des territoires avait indiqué rouvrir le dossier de la géographie prioritaire de la ruralité, précisant qu'il fallait se donner le temps d'y travailler. La définition d'une La définition d'une nouvelle géographie prioritaire des territoires ruraux est prévue à compter de 2021. Une mission inter-inspections a été lancée au début de 2020 pour faire un diagnostic et des propositions, mais ce chantier

rurale. Cet amendement reprend la préconisation du rapport sénatorial « Sauver les zones de revitalisation rurale (ZRR), un enjeu pour 2020 », présenté le 9 octobre 2019 par nos collègues Frédérique Espagnac, Bernard Delcros et Rémy Pointereau,

je vous remercie

Dans les discours, le Gouvernement, et le Premier ministre en particulier, ne cesse de se référer aux territoires. Alors, permettons à tous les territoires de notre pays de vivre, d'apporter leur richesse et de contribuer à la relance dont on parle tant. Faisons participer tout le monde

En effet, il est essentiel, pour obtenir un prêt, un taux intéressant et de meilleures conditions de remboursement, que la cotation Banque de France soit de bonne qualité.

60 % d'entre elles ne pourront pas reprendre leurs activités avant septembre, tandis qu'un quart ne pourront pas exécuter au moins 50 % de leur budget prévisionnel. Les associations employeuses sont particulièrement touchées, alors qu'elles emploient aujourd'hui 1,8 million de salariés. Afin d'aider le secteur associatif, le présent amendement vise à exonérer les associations employeuses de la taxe sur les salaires pour les rémunérations de 2020. Les associations qui payent de la taxe sur les salaires représentent environ 47 % des associations employeuses. Ce sont donc 74 000 associations qui pourraient être bénéficiaires Cette taxe représente aujourd'hui en moyenne 6 % de la masse salariale et 3,4 % du budget des associations, selon une étude du Mouvement associatif.

monsieur le rapporteur

Monsieur le rapporteur

Chez nous, l'essentiel de la fiscalité sur les entreprises repose non pas sur les bénéfices, mais sur les assiettes, en amont, c'est-à-dire qu'elle est déconnectée du résultat. Autrement dit, la fiscalité que supportent nos entreprises n'est pas liée à leurs performances économiques.

chance pour gagner la course ! Par ces impôts, nous laminons la compétitivité de nos entreprises, pour des produits à forte valeur ajoutée comme pour des produits plus basiques, tels que les masques de protection.

L'essentiel de ces impôts de production étant des impôts locaux, leur suppression reviendrait à restreindre les marges de manoeuvre fiscales des collectivités C'est pourquoi, monsieur le ministre, il faudrait approfondir en parallèle la question de l'autonomie fiscale des collectivités locales, en vue de les rendre à la fois plus libres et plus responsables.

et, dans le même temps, avoir des impôts de production trois fois plus élevés que ceux de l'Allemagne.

mais il ne s'agit pas seulement de la compétitivité du pays : il s'agit aussi du financement de la protection sociale. Si la C3S est un impôt de production particulièrement problématique, il faut alors trouver d'autres moyens

à prendre rendez-vous avec le Gouvernement, qui ne cesse de dire qu'il faut supprimer les impôts de production.

d'une recommandation de la Convention citoyenne pour le climat, vise à préciser le type d'entreprises concernées par le mécanisme de transparence et d'obligations environnementales prévu par cet article. Par souci de logique fiscale, il paraît plus pertinent de renvoyer aux entreprises ou groupes d'entreprises de plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est en effet le seuil retenu, au titre de l'impôt sur les sociétés, pour différencier, en particulier, le taux facial de prélèvement sur les bénéfices.

par voie de recapitalisation qu'elles prennent des engagements forts pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Cependant, cette exigence ne doit pas mettre en danger la survie des entreprises par des tâches et des contraintes supplémentaires. En l'occurrence, le seuil de chiffre d'affaires de 500 millions d'euros par la rédaction actuelle de l'article conduit à inclure une grande partie des entreprises de taille intermédiaire. Cet amendement vise donc à relever ce seuil afin de restreindre l'application de ces contraintes supplémentaires aux seules grandes entreprises, qui sont les mieux équipées pour mesurer et piloter leurs émissions de gaz à effet de serre. Il faut sauver les entreprises avant de chercher à toutes les verdir

Cet amendement vise à garantir une ambition suffisante des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui devront être pris par les entreprises concernées par l'obligation prévue par l'article 19, en fixant des objectifs minimaux de réduction par secteur d'activité.

d'une action de réduction des émissions, afin que les entreprises puissent être accompagnées pour établir leur reporting climat. Cet amendement est aussi une reprise d'une préconisation de la Convention citoyenne

ou, pour le moins, à une trajectoire de baisse des émissions qui soit conforme aux stratégies nationales bas carbone. L'article 19 vise donc à conditionner les prises de participation de l'Agence des participations de l'État au sein du capital des grandes entreprises à la souscription des derniers engagements forts en matière de transition écologique. Pour autant, cet article présente à nos yeux une lacune : il ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de ces engagements ; seule la non-présentation du rapport est sanctionnée.

en sorte que les grandes entreprises, en plus des pénalités précédemment énoncées, soient soumises à une interdiction de versement de dividendes. Cet amendement nous paraît indispensable : faute de sanction, nous n'obtiendrons pas un engagement total de ces entreprises dans la nécessaire transition écologique.

Cet amendement vise à améliorer explicitement la contrainte qui peut être exercée pour obtenir la publication des documents et informations mis en place.

alors qu'elle était en difficulté. Cette entreprise fait des bénéfices. Va-t-on la laisser verser des dividendes ? Va-t-on la laisser acquérir des actifs dans les paradis fiscaux ?

fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et des comptes publics. Il s'agit également d'exiger des sociétés bénéficiaires de respecter les dispositions de l'accord de Paris sur le climat et de remettre chaque année un rapport sur leur trajectoire de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, conformément aux dispositions du code de l'environnement, telles que renforcées par la loi Énergie-climat. Enfin, les entreprises soumises à la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre seront tenues d'avoir mis en oeuvre de manière effective un plan de vigilance. la solidarité nationale serait conditionnée à une responsabilité sociale, environnementale et fiscale des sociétés bénéficiaires. En restreignant le champ du dispositif aux seules entreprises dites moyennes et supérieures, nous tenons compte de la capacité des entreprises à faire face à ces obligations. Dans cette logique, l'amendement n'impose pas d'obligations pour les entreprises bénéficiaires du fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020, au regard des conditions d'éligibilité à celui-ci.

Il y aura des règles qu'il faut respecter. Si vous avez bénéficié de la trésorerie de l'État, vous ne pouvez pas verser de dividendes et vous ne pouvez pas racheter des actions », avait dit Bruno Le Maire.

Cet amendement vise à conditionner le bénéfice de l'ensemble des mesures d'urgence mises en place par l'État au respect des exigences de la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses

On sait que la première des mesures à prendre serait d'améliorer la liste des paradis fiscaux, mais on recule à chaque fois devant cette exigence. Dans l'immédiat, nous proposons de ne pas délivrer d'aides publiques aux entreprises qui déclarent des bénéfices dans les pays ayant des pratiques fiscales déloyales, notamment en termes d'impôt sur les sociétés.

La crise et la perspective de la destruction de près de 900 000 emplois en 2020, selon la Banque de France, rend largement caduque cette trajectoire financière. Il s'agit de tout remettre à plat, au vu de la situation actuelle.

pour les élections municipales, des élus ont fait valoir leurs efforts, en matière de gestion budgétaire, pour diminuer la pression fiscale exercée sur leurs administrés. Certains s'étaient même engagés de longue date sur une trajectoire de baisse des impôts, assortie d'une baisse des dépenses

M. Rémi Féraud. « Ceux qui payent aujourd'hui la taxe d'habitation pour lesquels on n'avait pas encore baissé, on peut peut-être attendre un peu plus d'années pour le faire parce qu'on est à un moment exceptionnel, parce que c'est assez légitime et que c'est au fond du bon sens. Voilà.

qui ne seront pas de trop dans les mois qui viennent. Par ailleurs, nous l'avons tous dit, l'actuelle crise sanitaire, économique et sociale a mis en grande difficulté

J'avoue notre incompréhension devant la cacophonie qui s'est installée dans l'exécutif ces derniers jours. Plusieurs engagements pris par le Gouvernement voilà deux ou trois jours n'étaient absolument pas

Nelly Tocqueville. Le présent amendement vise à reprendre le dispositif de 2010 relatif aux modalités d'attribution et de versement du FCTVA, afin de soutenir l'investissement public local.

et 2019 pourraient prendre en considération les dépenses afférentes à l'exercice précédent, à compter de 2021. Ainsi, pour l'année 2021, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2019 s'ajouteraient à celles qui sont afférentes à l'exercice 2020 pour le calcul des attributions du FCTVA.

alors que ces communes supportent des charges de centralité importantes. La perte de la fraction bourg-centre de la DSR menace aujourd'hui la pérennité des services de proximité qu'elles doivent assumer. En outre, ce plafonnement a engendré un effet de seuil extrêmement brutal, excluant une dizaine de communes du dispositif, dont plus de la moitié sont situées en zone de montagne. Il avait été convenu que ce sujet serait traité dans le cadre de la future réforme de la DGF

aux projets dont le coût n'excède pas 50 000 euros. Les subventions resteraient attribuées par le préfet de département.

pour une action ou un projet ayant été affecté par la crise actuelle. Cette demande s'inscrit dans la logique de la circulaire du Premier ministre relative aux adaptations des règles relatives aux subventions pendant la crise, qui permet aux pouvoirs publics de maintenir la totalité d'une subvention.

en part additionnelle à la fiscalité des ménages et des entreprises, avec, au fil du temps, un ajustement de cette part additionnelle, sans délibération des conseils municipaux ou du conseil syndical.

est de valoriser le recrutement d'étudiants de niveau mastère ou bac+5 en apprentissage, comme le préconisent la conférence des présidents d'université,

je vous présente les éléments de coordination suivants. Les crédits du budget général, hors remboursements et dégrèvements, sont augmentés de près de 600 millions d'euros, au travers de trois mesures. En premier lieu, une ouverture de crédits, à hauteur de 250 millions d'euros,

à tenir compte d'annonces du Gouvernement, notamment du plan de relance pour l'emploi des jeunes, qui inclut les contrats de professionnalisation dans l'aide exceptionnelle à l'apprentissage, ou des dispositions que nous venons d'examiner. En troisième lieu,

Ainsi, au terme de l'examen de ce projet de loi de finances rectificative, le solde budgétaire se dégraderait de près de 2,2 milliards d'euros par rapport au projet de loi déposé et le déficit s'établirait à 226,6 milliards d'euros.

Pour ma part, je suis très inquiet des sombres perspectives qui s'ouvrent pour notre pays. Je reste perplexe devant la stratégie suivie, cette fuite en avant budgétaire marquée par un un emballement du déficit et de l'endettement publics. Ainsi, après avoir épuisé le présent, on dévorera l'avenir, aurait sûrement dit le célèbre économiste Frédéric Bastiat. Avec un nouveau déficit de plus de 225 milliards d'euros, qui s'ajoute à une dette elle-même colossale, nous engageons notre responsabilité collective à l'égard des générations futures. Curieux paradoxe : j'entends de tous bords s'élever le mot « souveraineté », mais, « en même temps », nous nous plaçons entre les mains de créanciers étrangers. Aucun de nous, sur ces travées, ne peut s'exempter d'un examen de conscience. Il suffit de suivre le dérouleur des amendements pour constater que quelque chose ne va pas. La dépense paraît incontrôlée ; on injecte des crédits budgétaires comme on injecte un médicament qui soulage et permet de passer la nuit mais ne règle rien. Confrontée à sa pire récession depuis 1917, l'économie française est au bord de la débâcle. Pour financer tous les « plans Marshall », certains ont une solution : faire payer les riches. L'idée a pour elle la force de la simplicité, mais elle a les faiblesses de la démagogie, de la démagogie, celle qui consiste à voter contre le budget au motif qu'il ne serait jamais assez dépensier, comme on l'a vu à l'Assemblée nationale. L'issue serait la ruine pour tous ... D'autres cèdent au mirage de l'interventionnisme. Mus par une conception paternaliste de l'économie, ils croient pouvoir guider les comportements au travers de baisses ciblées de cotisations sociales et de fiscalité. À vouloir jouer au Meccano, on crée un monde de complexité qui entrave notre économie. ce chemin rendra la France dépendante d'autres pays plus agiles, plus performants. Par solidarité dans l'épreuve, je voterai ce texte, ... Ah ! ... mais je suis convaincu qu'une autre voie est possible. La France ne se redressera pas sans affronter ses propres faiblesses et sans revoir son fonctionnement en profondeur. Cela passe par la simplification de nos réglementations et de nos impôts. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.

sont pour le moment dans une grande incertitude et largement mises à contribution face à la crise, sans que nous sachions véritablement quelles seront leurs perspectives après 2020. Les deux

Je vais voter cet